Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

Hier, le président Bas, avec la cruauté délicieuse que nous lui connaissons, avait qualifié l'un des articles et ce texte en général de « tigre de papier ».

je veux bien que chacun ait sa liberté de parole et puisse dire tout ce qu'il souhaite, mais j'aime autant que les choses correspondent à la vérité. La vérité est celle que j'ai exprimée hier après-midi devant vous, à savoir que c'est sur mon initiative que j'ai proposé au président du Sénat ainsi qu'aux collègues

Je me permets, mes chers collègues, de vous dire que, lorsque je vous ai avertis de cela, vous m'avez dit que j'avais raison. Nous nous sommes donc organisés en conséquence, et pour cette raison-là, et, me semble-t-il, à la satisfaction de tout le monde. Sans autre forme d'arrière-pensées.

de loi visant à améliorer la trésorerie des associations dont la navette n'a pas encore abouti, est très bienvenue et attendue par le secteur associatif.

Il apparaît donc que l'article 12 A est satisfait et introduirait, qui plus est, une ambiguïté au regard des différences de forme qui peuvent exister entre les deux rédactions. Nous proposons donc de supprimer l'article 12 A.

Outre des précisions rédactionnelles, il a pour objet de renforcer l'effectivité du contrôle des financements étrangers prévus pour les associations au-delà d'un certain seuil, en permettant au préfet de saisir le juge afin qu'il puisse, si nécessaire, enjoindre aux associations de publier leurs comptes.

du mécénat plutôt qu'au sein de la loi de 1901, afin de ne pas créer de confusion sur le champ d'application du contrôle.

des ressources financières qui les alimentent. Les possibilités de contrôle des finances des associations doivent être étendues et améliorées, avec un focus tout particulier sur les ressources provenant des pays étrangers. Pour ce faire, l'état de ces fonds étrangers devrait faire l'objet d'un document à bien distinguer des comptes annuels des associations. À partir de ce document, le commissaire aux comptes effectuerait des attestations de type « ressources provenant de l'étranger » ou bien « avantages fournis par une personne étrangère

l'avis de la commission ? Ces deux amendements

Nous pensons que son apport est essentiel et, comme M. le sénateur l'a rappelé, la commission des lois a voulu renforcer l'effectivité de cet article en sanctionnant d'une amende de 9 000 euros le non-respect de l'obligation de publication des comptes. Renforcer

justifiant, ainsi, une obligation de déclaration à l'autorité administrative. De fait, il ne s'agit pas de viser tous les types de biens- meubles, immeubles, sommes d'argent, parts sociales ou prêts de main-d'oeuvre -sur lesquels peut porter l'opération juridique qui constituerait un avantage ou une ressource. Par ailleurs, nous souhaitons indiquer que les parts sociales ne constituent pas, en tant que telles, un avantage, puisque le don de parts sociales l'est et que les dons sont déjà bien mentionnés dans la liste. C'est donc une demande de retrait.

Hassani. La commission des lois a utilement aligné le régime de contrôle des financements étrangers des fonds de dotation sur celui qui est prévu par le projet de loi pour les associations loi 1901 bénéficiant de plus de 153 000 euros de dons. En continuité, ainsi que dans un souci de cohérence et de lisibilité, nous proposons d'opérer, au sein de l'article 12 relatif aux fonds de dotation, un renvoi aux dispositions de la loi de 1987 sur le mécénat, dans laquelle notre précédent amendement à l'article 12 visait à introduire des dispositions relatives au contrôle des financements étrangers des associations.

régies par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'en prévoit pas clairement l'accès en ligne. Cet amendement le précise. Quel est l'avis de la commission ? Favorable. Quel est

Le déploiement d'un registre numérisé des associations inscrites en Alsace-Moselle appelle des travaux sur ses contours. En revanche, il nous semble qu'une telle accessibilité en ligne de ces registres mériterait une expertise complémentaire à mener à la fois en lien avec les instances locales, mais aussi en interministériel. En effet, un registre des associations contient des données personnelles de ses membres. Il est, par conséquent, indispensable que nous puissions analyser la portée des données à rendre accessibles pour garantir le respect de la vie privée

La modernisation du registre des associations et associations coopératives d'Alsace et de Moselle, dont la tenue systématique sous forme électronique est prévue par cet article, ne prévoit pas la dématérialisation des formalités leur incombant. Pour le moment, toutes les démarches liées à la vie statutaire d'une association de droit local se font encore par courrier postal, ce qui crée une certaine iniquité entre les associations de droit local et les associations loi 1901. Or ces fonctionnalités étant particulièrement importantes pour les associations de droit local, cet amendement vise à leur mise en oeuvre effective.

La commission n'a pas adopté l'article 13, qui tend à rétablir un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au profit d'enfants qui ne bénéficieraient pas d'une réserve successorale en application d'une loi étrangère. À ses

des effets évidents dans le cadre des successions internationales soumises au droit anglo-saxon, alors que ces droits ne sont pas connus pour être discriminants envers les femmes. Toutefois, la commission a approuvé les articles 14 et 15, qui visent à renforcer la lutte contre la polygamie, naturellement, n'a pas sa place sur notre territoire. Nous affirmons clairement que vivre en état de polygamie en France doit faire obstacle au séjour. Dans le même esprit, nous proposons d'adopter un amendement de M. Roger Karoutchi, qui permettrait, en totale cohérence avec l'objet du projet de loi, de faire obstacle

La commission a précisé dans le texte que les professionnels de santé devraient expressément informer leurs patientes de l'interdiction de cette pratique. Elle a également adopté l'article 16 relatif au délit d'incitation et de contrainte à se soumettre à un examen de virginité, voté par les députés, pour poursuivre les « commanditaires »

visant toute personne qui procéderait à ces tests, et non pas les seuls professionnels de santé, étant précisé que les poursuites pour viol ou agression sexuelle devaient être privilégiées si les éléments constitutifs de ces infractions devaient être réunis. La commission a également conforté le dispositif de lutte contre l'excision en prévoyant une meilleure proportionnalité de la peine en cas d'incitation et de contrainte exercée sur une mineure pour qu'elle se soumette à ces mutilations sexuelles. Enfin, elle a renforcé le dispositif de signalement des mariages forcés ou frauduleux en prévoyant la constitution d'une base de données nationale recensant l'ensemble des décisions d'opposition et de sursis prononcées par le parquet,

non pas au dispositif proposé par le Gouvernement, mais au concept même de mécanisme réservataire. Les rapporteures y indiquent qu'elle porterait atteinte à la liberté individuelle et à la propriété privée, serait une entrave à la circulation de capital ou au développement de la philanthropie,

Sur ce dernier point, et sur le fait que les pays occidentaux ne connaîtraient pas d'inégalités entre les sexes lors des successions, il est heureux que les inégalités sociales entre les enfants puissent être résorbées par ce mécanisme. Sur l'égale protection entre les héritiers sur une partie de la succession, vous connaissez la position du groupe CRCE. Nous soutenons ces dispositions, qui constituent, certes, une entrave à la libre circulation du capital, mais, surtout, l'une des garanties possibles du respect de l'égalité entre les sexes. Le droit français ne vient pas s'immiscer de manière impudique dans la vie des familles. Au contraire, c'est parce que l'on connaît rarement l'intention d'un légataire, parce que « le testateur habile sait taire ou travestir la cause de sa préférence coupable » que la réserve héréditaire permet de ne pas s'encombrer de telle ou telle interprétation. L'égalité est proclamée sans interprétation. Elle est de droit et effective. En 2020, la Banque mondiale a mis à disposition un jeu de données qui met au jour que, dans 43 pays, les fils et les filles n'ont pas les mêmes droits de succession quand il s'agit d'hériter des biens de leurs parents. Dans 44 pays, les conjoints survivants n'ont pas les mêmes droits pour hériter des biens de leur époux décédé. Même si nous regrettons que cet article s'applique uniquement lorsque la loi étrangère ne prévoit aucun mécanisme réservataire, il constitue une avancée. Il faut le rétablir.

elle peut, par exemple, décider de tout laisser à son fils, et rien à sa fille, déshériter des enfants nés d'une précédente union ou des enfants dits « adultérins », etc. Ces enfants ne sont pas protégés. Le présent amendement vise non seulement à combler ce vide juridique, qui permet des discriminations potentielles, mais aussi à rendre la protection tout à fait concrète et effective. Grâce à cette disposition, l'enfant déshérité pourra récupérer sa part de réserve sur les biens situés en France

ne sont pas protégés par la réserve héréditaire : ils sont souvent déshérités sur le fondement de pratiques coutumières. Mesdames les rapporteures, je sais que vous craignez que la disposition ne s'applique aussi aux lois anglo-saxonnes, qui ne connaissent pas non plus la réserve héréditaire. Très sincèrement, je ne vois pas de raison de les en exclure

à l'enfant dans le besoin de réclamer une part de la succession. Ainsi, si l'enfant est déjà protégé dans les faits par le droit étranger, le droit de prélèvement ne jouera pas en France. Notre amendement tend en effet à préciser, contrairement à la rédaction initiale, que la loi étrangère ne doit permettre aucun mécanisme réservataire. Il autorise ainsi une appréciation concrète et factuelle de la loi étrangère, qui permet de vérifier si l'enfant est protégé ou non dans les cas d'espèce. Enfin, votre commission a supprimé l'obligation d'information renforcée des héritiers réservataires qui avait été mise à la charge du notaire. Le Gouvernement propose également de la rétablir, afin que les enfants puissent exercer leur droit en pleine connaissance de cause et à l'abri des pressions familiales. Nous considérons qu'il est inadmissible qu'en 2021, en France, des filles soient déshéritées parce qu'elles sont des filles et que certains veuillent appliquer des lois coutumières au mépris des lois de la République.

ce qui est soutenu par les auteurs de l'amendement n° 548 rectifié, n'a pas critiqué la réserve héréditaire en affirmant, en particulier, qu'elle nuisait à la circulation des capitaux

parce que nous contestons le bien-fondé de la réserve héréditaire, mais parce que nous avons estimé que les femmes étaient déjà protégées contre les discriminations les plus flagrantes imposées, par exemple, par la règle de tafadol, applicable dans la plupart des pays musulmans,

dans les successions soumises aux lois de pays de droit musulman, qui sont évidemment ceux qui sont visés par le texte, car, dans ces pays, la liberté successorale est très encadrée : c'est généralement la loi qui règle les successions.

ayant été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans sera systématiquement retiré par l'autorité administrative, sauf décision contraire dûment motivée. ? Cet amendement tend à prévoir le retrait systématique du titre de séjour pour l'étranger condamné à trois ans de prison,

Cela me semble assez normal ! Le présent amendement a pour objet de rendre automatique l'expulsion du territoire français d'un étranger qui ne respecterait pas cette disposition. Sinon s'installera une situation anarchique, en plus d'être immorale, favorisant un engrenage séparatiste. La polygamie est un état de vie contraire à notre droit. Elle occasionne par ailleurs de nombreuses situations de fraude aux prestations sociales. Il faudra réformer les organismes de la Caisse nationale d'allocations familiales pour que les contrôles des situations puissent être plus efficaces lorsque l'on soupçonne que des droits ont été indûment versés pour cause de polygamie. Difficile à constater tant la frontière avec la vie privée est ténue, la polygamie, dès qu'elle est avérée, doit faire l'objet d'un rejet sans concession. Il convient donc de prendre à bras-le-corps des décisions pour l'éradiquer. En ce bicentenaire de la mort de l'empereur, rendons un premier hommage à Napoléon I en combattant ceux qui piétinent sans vergogne son code civil ! Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement visant à l'expulsion des étrangers en situation de polygamie. Je suis certain

Nous siégeons dans cet hémicycle pour prendre des mesures, faire la loi, la modifier, l'inventer, la créer pour répondre à des situations nouvelles, même complexes

ne nous surprend pas de sa part. Il vise à renforcer la lutte contre le séparatisme en faisant obstacle à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour des individus dont il est établi qu'ils ont manifestement exprimé un rejet des valeurs de la République, ces principes mêmes que le titre du projet de loi dont nous débattons aujourd'hui appelle à protéger et qui justifient un renforcement des efforts dans la lutte contre la polygamie. Le Ceseda comprend déjà à divers endroits une réserve à la délivrance des titres de séjour, relative aux menaces pour l'ordre public. Les auteurs de cet amendement proposent très simplement de prolonger celle-ci en l'étendant aux situations des personnes ayant exprimé de manière indéniable leur rejet des principes républicains. Cela donnera aux autorités préfectorales et au juge les outils nécessaires pour agir dans les cas où une personne a, par ses actions ou par ses paroles, manifestement choisi de se désolidariser radicalement des valeurs de notre République.

partageons notamment l'absolue nécessité de défendre les principes et les valeurs de la République- c'est comme vous l'avez rappelé, madame la sénatrice, l'objet du présent projet de loi. Vous proposez d'introduire dans le Ceseda une disposition qui permette, au même titre que les menaces d'ordre public, une réserve à la délivrance du titre de séjour aux personnes qui ont exprimé leur rejet des principes républicains. Je veux d'abord dire que c'est ce que le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, et moi-même essayons de mettre

est un acte discrétionnaire : il ne peut pas être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt général, mais personne ne peut se prévaloir d'un droit à rester en France à l'expiration de son titre de séjour. Il s'agit ici de prévoir que, comme un motif d'ordre public, un rejet un rejet expressément formulé des principes de la République justifie le non-renouvellement d'un titre de séjour. C'est tout de même bien le moins. À cet égard, je regrette la tiédeur du Gouvernement, qui se borne

les femmes faisant l'objet d'un mariage polygame sont d'abord et avant tout des victimes. Nous pensons donc que l'Assemblée nationale a eu raison d'étendre le bénéfice du renouvellement automatique du titre de séjour, déjà prévu pour les personnes victimes de violences conjugales et familiales,

cette comparaison, il s'agit de montrer à quel point la pratique de la polygamie est minime. Si nous comprenons l'opposition qu'elle soulève à juste titre, nous ne saurions accepter que ce soit les femmes, principales victimes de cette pratique, qui en payent le prix. à revenir, et c'est là le problème, sur le renouvellement automatique de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à l'étrangère conjointe d'un Français polygame. Les auteurs de cet amendement

et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de reconnaître la polygamie comme une pratique subie par les femmes étrangères mariées de force et de leur accorder le renouvellement automatique de leur titre de séjour. La droite sénatoriale a supprimé en commission cet article au prétexte que le renouvellement automatique de la carte de séjour « vie privée et familiale pour les personnes victimes de pratiques de polygamie serait inopportun. En réalité, ce qui est inopportun, c'est le sort des femmes étrangères victimes de mariages forcés, qui perdent actuellement leur carte de résident lorsque leur mari est condamné pour polygamie. Cette double peine des femmes est inopportune. Nous refusons l'automaticité de la perte des titres de séjour. La polygamie constitue une oppression des femmes que nous jugeons intolérable dans la République. Dès lors, nous devons accueillir les victimes et les protéger plutôt que de les expulser. Tel était le sens de l'amendement de notre collègue Marie-George Buffet, que nous défendons ici, au Sénat. Quel

lorsque l'étranger a été victime de pratiques de polygamie. Dans ce cas, l'autorité administrative ne pourrait procéder au retrait du titre et devrait en accorder le renouvellement. C'est ce principe de renouvellement automatique que la commission des lois

ministre, devant la commission des lois du Sénat, vous avez affirmé : « Nous considérons donc que les pratiques dites " coutumières " telles que les mariages forcés, la polygamie, la discrimination en matière d'héritage et les certificats ou tests de virginité n'ont pas leur place en France. » Nous sommes également opposés à ces pratiques, car nous estimons qu'elles remettent en cause l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment le droit à disposer de son corps. Vous avez fait état, madame la ministre, de 200 000 femmes mariées de force sur le territoire national en 2020. Il convient donc non pas de sanctionner les femmes victimes de polygamie en les privant de la pension de réversion de leur mari, mais au contraire de s'attaquer véritablement au problème et de lutter contre la polygamie. Le texte ne prévoit aucune protection pour les femmes ayant épousé sous la contrainte un mari qui s'est avéré, par la suite, polygame. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel ? Cet amendement vise à supprimer l'article 15, qui tend à limiter de droit la réversion à un seul conjoint non divorcé. Ce dispositif est destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes les hommes et à faire prévaloir l'ordre public français. Il prévoit des garanties, il prend en compte les conjoints de bonne foi qui auront droit, dans tous les cas, à la pension.

de la polygamie. Il vise à préserver les droits de la première conjointe survivante en lui épargnant le partage de sa pension de réversion avec une autre femme mariée dans une situation de polygamie. Pour ce qui concerne les femmes ayant subi une situation de polygamie qu'elles ignoraient,

l'article 15 . En effet, à ses yeux, la polygamie est une situation matrimoniale qui n'est pas conforme à la législation française. La polygamie donne aux hommes tous les droits et aux femmes, tous les devoirs. La représentation nationale ne pouvait rester insensible à cet abus de vulnérabilité que constitue la polygamie de fait s'exerçant sur notre territoire. Malgré son interdiction, la polygamie continue d'exister dans notre pays, et il semble que les autorités et les pouvoirs publics français soient quelque peu impuissants à l'évaluer, à la contrôler, voire à la maîtriser. Les services de préfecture, qui sont en première ligne, sont bien en peine de fournir un chiffre quelconque quand on les interroge sur un phénomène qui leur échappe. Aussi Mme Boyer tient-elle à remercier la commission des lois d'avoir voté son amendement visant à introduire cet article 15 article 15 lequel prévoit expressément que les caisses d'allocations familiales avisent le procureur de la République de situations susceptibles de relever de cette infraction pénale. Les caisses d'allocations familiales ont alloué,

Les caisses d'allocations familiales (CAF) ne sont aucunement investies du rôle d'enquêter dans la vie intime et sexuelle des couples. Leur mission première est le versement de revenus, telles les prestations familiales ou les prestations sociales pour le compte de collectivités publiques, et la mise en oeuvre d'une action sociale destinée aux allocataires. telle intrusion dans la vie intime des familles par un organisme comme la caisse d'allocations familiales est liberticide. Elle porterait une atteinte manifeste aux principes de notre République que ce projet de loi prétend renforcer. comme toutes les sociétés démocratiques en Europe, est tenue au respect de la vie privée et familiale des individus, comme le prévoient les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cette injonction faite à certaines jeunes filles est une véritable violence que nous ne pouvons que dénoncer. C'est bien de violence qu'on parle : une violence psychologique, une pression insupportable, qui alimente la peur chez de nombreuses jeunes filles, y compris de représailles. Les témoignages de professionnels, dont celui de Ghada Hatem, gynécologue et fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, sont très éclairants. Elle explique très bien que délivrer ces certificats, sans bien évidemment pratiquer de tests, peut sauver la vie de jeunes femmes. En outre, les médecins peuvent s'appuyer sur l'Ordre des médecins, qui interdit déjà cette pratique, pour entamer un dialogue. Prévoir dans la loi l'interdiction de ces certificats, avec pénalisation des praticiennes et des praticiens, risque d'avoir plusieurs effets pervers. Cela pourra mettre à mal un lien qui se crée entre la jeune fille et le professionnel, permettant d'évoquer d'autres problèmes plus larges : l'intimité, la prévention et la santé sexuelle.

ne soyons pas naïfs ! Il y aura des contournements de cette interdiction, même si j'ai bien noté que l'article 16 vise à pénaliser la réalisation d'examens. Je crains le développement de filières clandestines sur lesquelles nous aurons du mal à avoir une visibilité ou une maîtrise. Sur des sujets aussi sensibles, il nous faut écouter les professionnels. Personne ne réclame l'inscription dans la loi d'une pratique déjà interdite par ailleurs. Surtout, tout le monde dénonce la pénalisation des médecins.

Quelle inversion des valeurs ! Que se produira-t-il quand la jeune fille rentrera chez elle avec sa petite enveloppe et son petit certificat de virginité à l'intérieur ? Elle épousera une personne qui a choisi comme acte fondateur du mariage,

une personne qui a exigé un tel certificat. Elle sera donc aux prises avec des pressions terribles. On peut gager que sa dignité de femme ne sera pas particulièrement respectée le reste de sa vie, s'il a fallu ce petit papier, ce certificat de virginité. Je préfère que la République soit courageuse et qu'elle dise clairement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Dans la République française, je souhaite donc que les certificats de virginité ne soient pas permis.

: La parole est à Mme Marie-Pierre Monier. En commission des lois, les socialistes ont soutenu l'interdiction d'établir un certificat de virginité. Un amendement visant à renforcer l'information de la jeune fille ou femme a été en partie adopté. obligent le professionnel de santé à informer la patiente concernée de l'interdiction de cette pratique. Nous souhaitons néanmoins compléter la protection que notre société doit à ces femmes contraintes par leur entourage de se soumettre à ces pratiques visant à établir leur virginité. Selon nous, l'accompagnement doit inclure également l'orientation de la femme vers les organismes judiciaires et associatifs spécialisés. Le seul rappel de l'interdiction n'est pas de nature à protéger suffisamment la jeune femme des risques qu'elle encourt. L'approche complémentaire des organismes associatifs ou judiciaires permet de déconstruire l'exigence de virginité et les présupposés patriarcaux que nous combattons.

a des ressources, qu'elle peut s'en sortir sans cela, je refuse de délivrer ce certificat. Je lui fais de la pédagogie, je lui parle des droits des femmes, des combats des générations précédentes pour que les femmes puissent disposer de leur corps. Mais dans certains cas, pour les très jeunes femmes notamment, ma priorité est d'abord de les protéger. Et si la délivrance d'un certificat de virginité est le seul moyen, je le fais et je l'assume. » Elle évoque aussi les dangers qui pèsent sur ces jeunes femmes, qui peuvent être renvoyées au bled

? Il nous semble absolument fondamental qu'un document soit remis afin que cette jeune femme soit protégée si elle ne revient pas avec le certificat attendu par sa famille. Car, très souvent, ce n'est pas elle qui demande ce document,

important de prévoir un dispositif complet. Ce n'est pas du bavardage. Puisque la France décide d'inscrire dans son droit l'interdiction de cette pratique, il faut que la jeune femme puisse vraiment s'en prévaloir, y compris auprès de ceux qui, dans sa famille, lui demandent

les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ». Il dispose également : « Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire [ ...]. » Cette disposition, introduite par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, est à saluer. Elle est cependant insuffisante, notamment pour protéger les femmes majeures. Dans une étude du réalisée en 2019 auprès de 431 participants, 29 % des médecins interrogés ont affirmé avoir déjà été sollicités pour délivrer un certificat de virginité. Ces professionnels de santé ont rapporté que, dans bien des cas, cette demande n'émanait aucunement de la patiente, mais de son futur conjoint, de la famille de la patiente ou de la future belle-famille de celle-ci. Les phénomènes d'emprise et de pression sociale dans ces situations ne sauraient être négligés. Étant sous influence, la patiente n'est souvent pas en mesure de consentir à ce que son médecin alerte le procureur de la République, sans pour autant qu'elle soit considérée en « incapacité physique ou psychique », comme cela est prévu à l'article 226-14 du code pénal. Conscient de l'ascendant que peut avoir l'entourage de sa patiente sur celle-ci, le professionnel de santé doit pouvoir lui porter secours en toute circonstance. Le présent amendement vise donc à faire des professionnels de santé des lanceurs d'alerte, en leur permettant de saisir le procureur de la République lorsqu'il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d'attester la virginité d'une femme. Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra prendre des mesures de protection au bénéfice de la femme, mener une enquête et diligenter d'éventuelles poursuites à l'encontre de ceux qui ont été à l'initiative de la demande du certificat de virginité.

ministre. Madame, vous êtes simpliste : pour vous, le monde, c'est oui ou non ! Cela ne marche pas comme ça

Cependant, lesdits certificats de virginité ne sont pas, pour la plupart, délivrés par des professionnels de santé. La réalité de notre pays tiers-mondisé oblige à élargir le dispositif prévu par ce projet de loi. Aujourd'hui, en France, des pseudo-médecins, des usurpateurs de titres officiels ou des référents communautaires, comme des figures cultuelles, sont sollicités pour attester de la virginité d'une personne avec ou contre son gré. On entend peu les pseudo-féministes autoproclamées, adeptes des combats idéologiques, comme l'écriture inclusive, sur ces sujets qui sont une réalité dans notre pays La dignité des femmes est pourtant bafouée par l'établissement de tels certificats, que l'on n'exige jamais des hommes. C'est la culture exogène de l'islamisme importé par l'immigration sur notre sol, contraire à nos modes de vie, qui fait des femmes des suspectes. Il est loin l'amour courtois de notre belle culture française Le présent amendement prévoit que la simple délivrance des certificats constitue un acte de faux, par lequel un individu, même non professionnel, commet un double délit consistant, d'une part, à établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, et, d'autre part, à faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Or ces délits sont répréhensibles, aux termes de l'article 441-7 du code pénal. Il faut mettre un terme à ces pratiques communautaristes étrangères en inscrivant, par la voie de cet amendement que je vous invite à adopter, un interdit clair, pour un professionnel ou un

Marie-Pierre Monier. L'Assemblée nationale a créé un nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique, qui pénalise l'examen visant à établir la virginité. Il assimile cet examen à un viol s'il a donné lieu à pénétration ou à agression sexuelle. Les rapporteures de la commission des lois ont écarté cette qualification pénale pour des motivations qui nous posent problème. Il a notamment été rappelé que l'élément constitutif de l'acte par violence, contrainte, menace ou surprise, ne pouvait être établi, du fait du consentement de la jeune fille ou de la femme. Selon nous, il n'est pas envisageable d'interroger le consentement d'une personne qui a grandi, qui a été éduquée, et dont l'avenir dépend de la soumission à des pratiques culturelles et à des normes sociales familiales. La jeune femme se trouvant dans cette situation est dans une position d'emprise telle qu'elle ne peut que consentir à ces rites. Parfois même, il arrive que certaines femmes consentent à un mariage forcé pour quitter le carcan familial, et pour retrouver un nouveau carcan conjugal guère plus permissif. Nous souhaitons que l'on cesse d'interroger le libre arbitre de ces jeunes femmes. L'assimilation de l'examen de virginité à un viol ou à une agression sexuelle revient à formaliser l'interdit clair de cette pratique rétrograde.

La solution proposée par la commission est juridiquement plus robuste et plus large puisque seraient concernés les professionnels comme les non-professionnels. En effet, si l'examen de virginité est considéré comme illégitime- et même moyenâgeux, selon moi -, alors la différence de traitement entre les professionnels et les non-professionnels n'est pas fondée et constitue une rupture d'égalité. Une lecture pourrait même conduire à ne pas pouvoir poursuivre pour viol ou agression sexuelle un médecin qui procéderait à des examens d'ordre gynécologique sans aucun motif médical. Cela n'empêcherait pas les médecins de vérifier si l'hymen d'une victime d'agression sexuelle a été rompu, l'examen visant alors à attester des violences subies. La solution que la commission propose est la suivante. Un médecin ou un non-médecin qui pratique un test de virginité sur une jeune fille obligée de s'y soumettre par son entourage commet un viol ou une agression sexuelle, selon qu'il y a ou non pénétration, en en application du droit existant- il n'y a pas besoin de changer la loi. Un médecin ou non-médecin qui pratique un examen de virginité sur une jeune fille qui s'y soumet sans pression de son entourage ni menace ni violence est coupable du nouveau délit créé à l'article 16 , que j'ai déjà évoqué, des peines fortes de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, la peine étant aggravée si c'est une mineure. À aucun moment, nous n'avons soutenu que « la victime à qui l'on somme d'attester de sa virginité pourrait consentir à un tel examen ». Si elle est contrainte, alors c'est un viol ou une agression sexuelle et les dispositions du code pénal

Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n'étant pas accompagnés du titulaire de l'autorité parentale doivent disposer d'une autorisation. L'objet de cet amendement est d'adjoindre à cette autorisation un certificat de non-excision pour tout enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale. Un décret du Conseil d'État pourrait déterminer les conditions d'application de cette disposition. Il conviendrait également d'envisager un examen médical avant le départ et dès le retour de l'enfant mineur sur le territoire français. Ainsi, si le médecin ne constate aucune mutilation, le certificat pourrait être remis aux représentants légaux de la mineure ; si,, le médecin constate une mutilation, le certificat sera directement transmis

à M. Stéphane Le Rudulier. Dans certaines maternités, des équipes médico-chirurgicales se sont mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de mutilations comme l'excision. Ces initiatives permettent d'accompagner et de sensibiliser les patientes en abordant tous les aspects de prévention, de conseil, de soutien et d'information, avec un rappel du cadre législatif français. français. Lorsqu'un médecin ou une sage-femme constate à l'occasion d'un examen médical qu'une parturiente a subi une mutilation de nature sexuelle, le praticien de santé devrait pouvoir remettre à celle-ci une « charte de protection de de l'intégrité génitale de la femme ». Ce document présenterait le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l'interdiction de toute forme de mutilation prévue par le code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l'occasion d'une mutilation génitale. Quel l'avis de la commission ?

à M. Stéphane Le Rudulier. Le carnet de santé est un document qui contient les éléments d'information médicale nécessaires au suivi de la santé de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Son utilisation est réservée aux professionnels de santé et sa consultation soumise à l'accord des parents. En tant que document officiel soumis au secret professionnel, il est un outil de liaison entre les différents agents du milieu médical.

contrairement à ce qui a pu être indiqué précédemment. Ce message rappellerait, dans un premier temps, les risques de ces pratiques sur l'intégrité physique et psychique de l'enfant et, dans un second temps, la sanction prévue par le code pénal. Ainsi, le service de protection maternelle infantile du département de la Seine-Saint-Denis prévoit déjà que, dans le cadre de la mission de protection infantile, les familles sont systématiquement informées de manière individuelle ou collective de la gravité des mutilations, de leurs conséquences sur la santé et de leur caractère illégal.

il y a eu le plus grand nombre de poursuites pénales pour des faits de mutilations sexuelles : environ 29 procès depuis 1979.

du Gouvernement ? J'associe le Gouvernement, si Mme la rapporteure me le permet, à l'hommage qu'elle vient de rendre à celles qui se sont battues pour interdire l'excision et les mutilations génitales. Je voudrais vous rappeler que le Gouvernement a lancé, avec le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, il y a un an et demi de cela, un grand plan contre l'excision, doté de moyens. Nous avons, par exemple, multiplié par trois la subvention de l'association Excision, parlons-en ! et avons décidé de financer davantage la Fédération GAMS que j'évoquais précédemment. Par ailleurs, nous avons également lancé une étude de prévalence

La commission des lois a supprimé l'article 16 A adopté par l'Assemblée nationale,

Pour notre groupe, la sensibilisation des enseignants à l'excision et aux mutilations sexuelles féminines est extrêmement importante. Ce problème,

adaptée des enseignants qui peuvent aider à la détection et, donc, à la protection des jeunes filles, et faire en quelque sorte de la prévention. En France, plus de 60 000 jeunes filles sont concernées par des mutilations sexuelles génitales. Notre Haute Assemblée a

avec Hadja Idrissa Bah, qui était alors présidente du Parlement des enfants de Guinée, et Annick Billon, présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Ne pas vouloir ajouter ces précisions dans la loi nous semble contradictoire avec la volonté affichée par le Sénat

cela ne va pas de soi -que l'existence des mutations génitales et sexuelles fait partie de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et, d'autre part, d'inciter à faire appel à des associations

précise : « Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. »

le constat de cette lacune avait fait l'objet d'un large consensus sur les travées du Sénat, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Ainsi, il nous paraît essentiel de réaffirmer que ces séances annuelles d'éducation à la sexualité doivent bien avoir lieu, car ces cours présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes, contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et constituent, de ce fait, un outil pédagogique et préventif précieux pour faire vivre ces principes de la République

qui a la responsabilité de ces séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, fait valoir que l'éducation peut être abordée en SVT, mais qu'elle peut également se déployer lors d'échanges ayant lieu en dehors des temps d'apprentissage,

de l'emprise de l'entourage, qui la place en situation de grande vulnérabilité. En conséquence, cet amendement tend à supprimer les alinéas relatifs à l'infraction lorsque la victime est d'accord pour subir un tel examen.

enregistrés à l'état civil français par la représentation diplomatique ou consulaire française territorialement compétente. En effet, la transcription, en droit français, du mariage d'une personne française avec une personne étrangère, célébré par une autorité étrangère légitime pour le faire, produit des effets civils en France, pour les enfants et les époux, en permettant notamment d'obtenir la nationalité française. Étant donné que la demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente, en fonction du lieu de célébration du mariage, il revient à cette même autorité de prendre des mesures de prévention nécessaires pour empêcher, au maximum, la transcription de mariages dont l'objet serait d'obtenir la nationalité française sans reposer sur le consentement réel, sérieux et intègre qu'exige l'article 146 du code civil. Ces fraudes, qui permettent la célébration de mariages simulés, que les deux conjoints soient au courant ou non, ouvrent la porte à une immigration clandestine légalisée et sont la cause de l'explosion des statistiques d'annulations de mariage. L'obtention de la nationalité par le mariage est la première cause de l'immigration en France ; il faut la contrôler. Notre droit doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour empêcher les nombreuses fraudes. La nationalité française s'hérite ou se mérite ; elle n'est pas une coquille vide et ne doit pas se laisser violer. L'officier de l'état civil doit donc faire réaliser une audition commune ou des entretiens individuels avant la transcription du mariage célébré par une autorité étrangère, afin d'éviter toute tentative de fraude à la nationalité française. Tel est le sens de cet amendement, que je vous propose, mes chers

à M. Stéphane Le Rudulier. Les officiers d'état civil doivent obligatoirement procéder à l'audition des futurs époux, préalablement à la publication des bans, afin de détecter le défaut d'intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.

de vérifier que le mariage envisagé n'est ni forcé ni frauduleux. Dans les cas où il existe des doutes sérieux quant à la sincérité d'un mariage, cet officier doit saisir le procureur de la République. Il est nécessaire que la décision de ce dernier intervienne dans un délai rapide, au regard de l'urgence de la situation,

Le projet de loi instaurait un questionnaire unique pour tous les maires ; c'est très bien, mais cela soulève la question de l'adaptation de ceux qui qui sont interrogés lors des entretiens individuels, donc cela suppose que le questionnaire change très régulièrement. De la même manière, il s'agit ici d'une question de mise en oeuvre. Je serai plus insistant que Mme la rapporteure, qui a dit les choses en termes très mesurés

prévoir tous les échanges d'un officier d'état civil avec l'un des mariés. Un questionnaire ne peut être qu'un document qui oriente une discussion

il convient d'obliger le ministère public, saisi par le maire, à surseoir automatiquement à la célébration d'une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier d'état civil et aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder

Enfin, le pouvoir d'appréciation du procureur de la République est une condition de la constitutionnalité du dispositif de contrôle préalable de la validité des mariages. Il nous semble impossible de le supprimer.

importants. Nous invitons le Sénat à prendre en considération les difficultés que les communes rencontreraient pour supporter les contraintes qu'impliquerait une telle réforme. Nous relevons que cet amendement vise à apporter une certaine souplesse au dispositif de consultation, en ce que ce que celle-ci pourrait également être effectuée par les procureurs de la République. Toutefois, dans les faits, ces dispositions ne pourraient pas être appliquées avant plusieurs années au moins, faute pour les procureurs de la République de disposer

Mme Esther Benbassa. Si ce projet de loi entend réellement réaffirmer les principes de la République, au premier rang desquels le principe de laïcité, il ne saurait être uniquement le symbole de la stigmatisation gratuite d'une certaine partie de la population française, notamment des musulmans. Au contraire, il devrait être vecteur de progrès sociétaux, en l'occurrence en matière de droit des femmes. Souvenons-nous de quelques errements de la jurisprudence,

à disposer de leur corps et à vivre librement leur sexualité. Pour tenter d'abréger ce long chemin, le présent à amendement vise à exclure la virginité des époux du champ des qualités essentielles pouvant justifier une annulation du mariage au sens de l'article 180 du code civil. Cette précision n'est aucunement superfétatoire,

Le droit fondamental au mariage et reconnu par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour autant, il existe déjà des conditions au mariage : des conditions de fond- âge minimum,

la régularité de séjour, mes chers collègues. En tout cas, nous devrions empêcher l'accès à la nationalité française par le mariage ou la limiter davantage.

Mme la rapporteure.

très clairement, en indiquant que le caractère irrégulier du séjour ne permettait pas de s'opposer au mariage, car ce dernier constitue une liberté fondamentale.

me choque quelque peu, surtout si c'est sujet à caution pour une régularisation. Adopter cet amendement, ce serait aussi saisir officiellement le Conseil constitutionnel pour qu'il se positionne de manière très claire, au-delà de la jurisprudence, sur les cas d'espèce qu'il a pu rencontrer.

Toutefois, l'article R. 2122-10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil. Aux termes de

mariages frauduleux. Ces référents seraient chargés de conseiller les autres officiers d'état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans un but autre que l'union matrimoniale. Cela permettrait d'accroître l'expertise requise en cas de doute,

Nous avons eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises au cours de nos débats sur ce texte : oui, l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe républicain. Il est essentiel de le faire vivre dans l'ensemble de nos territoires et de le décliner au premier échelon démocratique, celui des 35 000 communes. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux la création de ces conseillers municipaux dédiés, qui constitueront des interlocuteurs privilégiés sur l'ensemble des questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, au sein de chaque commune. Si les mariages forcés ont constitué le point de départ de notre réflexion, les officiers d'état civil ayant fait état d'un manque de formation et de sensibilisation

C'est particulièrement le cas en milieu rural. Dans ces territoires où sont commis la moitié des féminicides- 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural ! -, les élus constituent parfois le premier maillon de la chaîne de prise en charge, faute d'autres structures vers lesquelles se tourner. Ils pourraient dans ce contexte trouver l'appui nécessaire auprès d'un tel correspondant, désigné à l'échelon de la collectivité. Soutenus dans leur action par le réseau des directions régionales et les délégués départementaux aux droits des femmes et à l'égalité, ces correspondants contribueraient à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans l'ensemble de nos territoires en centralisant et en relayant activement l'ensemble des informations liées à ces thématiques, ainsi que les initiatives locales auprès du conseil municipal et des habitants de leur commune.